La promotion des marchés financiers dans un espace déréglementé et sans frontières – pour le capital –, notamment en Europe, scelle le passage du régime économique d’après guerre à l’économie financiarisée contemporaine. » La liquidité L’impératif de liquidité ! Voilà qui légitime l’accumulation primitive de capital issue de marchés autorégulés avec une possibilité infinie d’échanges, à tout moment et désormais à l’échelle de

faisant perdre de vue l’objectif même de la finance de marché : le financement de l’économie productive et, consubstantiellement, des États, par la mise en relation entre un épargnant et une entité publique ou privée.

roulent maintenant pour des multinationales de la spéculation, dont le sens des affaires n’a que peu d’égards pour la production ou l’économie réelle et encore moins pour les travailleurs – des obstacles, tout au plus…

! –, que l’on échange et sur lequel on spécule. Les marchés alternatifs sont régis par des règles de transparence et d’équité moins exigeantes, si bien que les plus gros opérateurs de marchés peuvent s’échanger un titre en une nanoseconde, bénéficiant ainsi des écarts de cotation entre les marchés réglementés et les marchés alternatifs. Dans chacune des failles se glisse un appétit, une prédation. Loin d’être des effets de bords d’une politique publique de régulation, ces failles correspondent précisément à l’intention des libéraux européens et nationaux : plus d’échanges de capitaux, à n’importe quelles conditions, pourvu que le système tienne jusqu’à la prochaine folie, jusqu’à la prochaine crise… la confiance, dopamine des marchés, ne mérite aucun commentaire : « se dit de l’assurance qu’on prend sur la probité, sur la discrétion de quelqu’un ou de quelque chose.

Euronext, qui doit son existence à la fusion des bourses belge, néerlandaise et française, rejointes depuis lors par quatre places boursières supplémentaires, est un opérateur de bourse paneuropéen lui même coté sur le marché français. Euronext, c’est 513 millions d’euros de bénéfice en 2023 – un record –, 1 900 émetteurs et 6 600 milliards d’euros de capitalisation boursière.

L’attractivité de la place financière française est secouée par l’annonce récente d’un éventuel transfert de la cotation principale de TotalEnergies vers les États Unis. Les liquidités y seraient abondantes pour les entreprises pétrolières, quand nous préférions, de ce côté ci de l’Atlantique, les énergies renouvelables.

Paris est déjà le premier marché boursier européen du point de vue de la capitalisation boursière, devant Londres. Les marchés se portent bien, les entreprises cotées tout autant. Nul besoin, donc, de légiférer en ce sens. D’ailleurs certaines dispositions du texte sont même contre productives ; nous proposerons de les supprimer.

le 8 janvier 2024, le Gouvernement annonçait l’arrivée au printemps suivant d’un texte sur l’attractivité financière de la France. Finalement, le choix a été fait de passer par une initiative parlementaire, qui permet d’éviter la production d’une étude d’impact et l’avis du Conseil d’État.

mais également à la défense, à l’heure où le monde se réarme, ou encore à la transition numérique de nos entreprises. Ce texte part d’un constat clair : les financements bancaires peinent à satisfaire, en France et en Europe, les besoins des entreprises et les projets de financement public tendent à devenir particulièrement restreints. Pour remédier à cette situation, l’auteur de la proposition de loi et le Gouvernement font valoir leur volonté de faire appel au financement de marché.

La pression pour l’obtention de résultats financiers ou la perte de contrôle sur les choix stratégiques peuvent entrer en contradiction avec d’autres objectifs auxquelles sont attachées nos entreprises.

Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, heures avant nos débats d’aujourd’hui, la septième édition du sommet Choose France réunissait plus de 180 chefs d’entreprise étrangère à Versailles,… Royal ! … avec, à la clé, une excellente nouvelle pour notre économie : plus de 15 milliards d’euros d’investissement dans 56 nouveaux projets. projets. C’est tout simplement un nouveau record, et, comme tous les records, celui ci est fait pour être dépassé : nous pouvons aller encore plus loin dans le renforcement du financement des entreprises et de l’attractivité de la France. Loin d’être une lubie financière, l’attractivité de notre pays est une réalité palpable, dont les effets se font ressentir sur notre économie. Vous l’avez dit, monsieur le ministre, si les annonces se sont faites dans un château, les parpaings, eux, sont posés partout en France, et si notre pays est aujourd’hui en tête du classement européen des investissements étrangers, ce n’est pas dû au hasard. Il faut certes reconnaître que l’Allemagne souffre davantage que nous de la guerre en Ukraine et que les Britanniques subissent encore les nombreuses conséquences du Brexit, mais le travail accompli depuis 2017 n’est pas étranger aux résultats positifs que nous enregistrons en matière d’attractivité. Bien au contraire, ces résultats sont le fruit d’un travail de longue haleine et des réformes menées par la majorité Les réformes liées à la fiscalité, au foncier, au prix de l’électricité, au marché du travail, ainsi que la création du prélèvement forfaitaire unique et la dynamisation de notre tissu entrepreneurial au travers de la loi Pacte sont à l’origine de ces succès.

Force est de constater que la majorité des banques anglo saxonnes ont choisi d’établir leurs activités de marché à Paris. Depuis 2021, cela représente plus de 5 500 emplois bancaires et financiers. J’ajoute que de nouvelles banques internationales s’installent actuellement à Paris, comme la banque émiratie First Abu Dhabi Bank et la banque nigériane Zenith Bank, sans oublier le nouveau campus européen de la banque américaine américaine Morgan Stanley, inauguré lundi dernier, qui créera 100 emplois supplémentaires, essentiellement des financiers et des chercheurs. Toutefois, en prenant du recul, on se rend compte que le secteur financier contribue de manière considérable à la prospérité économique de notre pays. Les données chiffrées sont éloquentes. Selon les chiffres de Paris Europlace, en Île de France, plus de 20 000 nouveaux emplois directs et indirects ont été créés entre 2017 et 2022. À l’échelle du pays, en 2023, quelque 1 815 décisions d’investissement international ont été recensées, permettant la création ou le maintien de quelque 60 000 emplois à horizon de 2026. Ce sont des investissements qui bénéficient à l’ensemble du territoire, puisque 49 % des projets sont réalisés dans des communes de moins de 20 000 habitants, à l’image de l’installation du futur centre de données de Microsoft dans le village de Petit Landau, dans le Haut Rhin. Le site est censé fonctionner uniquement à partir d’énergies renouvelables et devrait permettre,, de créer 200 emplois.

200 emplois sont promis, ainsi que 300 millions d’euros d’investissement dans un secteur clé, celui de la fabrication des batteries de véhicules électriques. Pensons encore à l’usine aéronautique de la société Lilium, destinée à la conception d’avions électriques, dont l’entrée en service est prévue pour 2026, quelque part en Nouvelle Aquitaine, avec 850 emplois à la clé. Voilà autant d’exemples d’investissements et de projets dans tous les territoires, avec un objectif très clair : que la France puisse redevenir une puissance industrielle. Renforcer l’attractivité de la France n’est donc pas qu’un slogan, c’est un cap politique et stratégique. Au delà des créations d’emplois, ces investissements jouent dès à présent un rôle décisif dans le plein emploi et donc dans le désendettement de la France. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons renforcer le financement des entreprises et l’attractivité de notre pays, grâce aux mesures qui sont présentées dans ce texte. Nous devons permettre à nos entreprises d’être encore plus compétitives et de s’adapter aux évolutions technologiques. Comment

Ensuite, le texte vise à soutenir la compétitivité des entreprises françaises dans leurs échanges internationaux, grâce à la reconnaissance des titres transférables électroniques, à leur définition juridique et à la reconnaissance Plus de 20 % des flux du commerce extérieur français sont adossés à ces titres transférables, ce qui n’est pas négligeable. Enfin, le texte contient des mesures qui adapteront notre droit interne aux nouvelles réalités du secteur, afin, là encore, de renforcer l’attractivité de notre législation. Concrètement, l’article 10 facilitera par exemple la numérisation des réunions pour les organes des sociétés commerciales, quand l’article 11 permettra à la cour d’appel de Paris de se spécialiser dans l’arbitrage international. Mes chers collègues, toutes les mesures que je viens de citer sont nécessaires pour renforcer notre attractivité. Pour séduire toujours plus d’investisseurs étrangers, il nous faut gagner en agilité et adapter notre arsenal juridique. Si notre savoir faire et nos formations permettent à notre pays d’être encore un formidable vivier de talents, nous ne devons pas nous empêcher d’attirer ceux qui sont venus d’ailleurs, avec toutes les conséquences positives que cela peut avoir sur notre économie et notre industrie. Nos concitoyens et les élus locaux le savent pertinemment : derrière une France plus attractive se cache en réalité une mosaïque de territoires qui peuvent en tirer parti.

Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs,

? Ce texte serait justifié par ses effets attendus en matière de création d’emplois, de rentrées fiscales et d’amélioration de la balance des paiements, mais rien ne le démontre.

Il est possible que, censé faciliter la croissance des start up en favorisant les levées de fonds, ce texte produise en réalité l’effet inverse : des entreprises de plus grande taille pourraient bénéficier du dispositif au détriment des start up. Le

Même en matière de droit du travail et de modalités de licenciement, votre approche est un alignement libéral vers le bas, monsieur le ministre. Vous me direz qu’il s’agit de traders très bien payés, mais pourquoi enfoncer encore un coin dans notre droit du travail ? Est ce vraiment le moment ?

des entreprises aux marchés financiers n’est pas spécifique à la France, puisque, dans son rapport remis au Gouvernement au mois d’avril dernier, Christian Noyer relève que ce problème est généralisé en Europe : notre continent exporte son épargne vers des produits de taux étrangers et importe des capitaux du reste du monde pour financer en fonds propres le développement à long terme de ses entreprises.

Cette proposition de loi souffre également d’un manque de fondement. Aucune étude d’impact ne vient étayer son potentiel intérêt ou ses éventuels effets délétères : dès lors, comment le législateur pourrait il travailler en connaissance de cause ? sur le fond, vous nous demandez d’approuver un texte de financiarisation de notre économie réelle. Si nous ne nions pas les problématiques de l’investissement productif et de son financement, nous défendons, pour notre part, le financement de proximité des entreprises.

Si cette proposition de loi part d’intentions louables, la copie rendue n’est réellement ni convaincante ni suffisante. Simplification administrative, facilitation du financement public et privé des investissements,

européens. La compétition internationale n’a jamais été si féroce : il faut se battre pour rester en tête et chercher, encore et toujours, à améliorer ses performances. En effet, à chaque investissement réalisé, ce sont des emplois qui sont créés, des technologies qui se développent et des territoires qui retrouvent des couleurs. Ce sont aussi – ne le perdons pas de vue – des recettes fiscales à venir.

Si le Président de la République peut convaincre des dirigeants étrangers à Versailles, c’est aussi et surtout parce qu’un travail collectif a été mené : réforme du marché du travail, baisse de l’impôt sur les sociétés et des impôts de production, réforme des retraites et de l’assurance chômage. Mais – j’y insiste – la compétition internationale n’a jamais été si rude. Les tensions géopolitiques sont à leur comble. Il faut poursuivre le travail pour préserver la compétitivité de notre pays et donc son attractivité : il y va de l’avenir de notre modèle social, de l’avenir de notre jeunesse tout entière. En ce sens, nous devons aussi aider nos jeunes entrepreneurs.

notre groupe accueillent très favorablement cette proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. Pour l’essentiel très technique, permettra de moderniser certaines dispositions de notre droit devenues désuètes. Mes chers collègues, préserver la compétitivité de nos entreprises, c’est aussi garantir un cadre législatif en phase avec les pratiques des entreprises et des investisseurs.

et, surtout, soutenir nos PME. Miser sur l’innovation technologique et sur l’initiative individuelle, c’est enclencher le cercle vertueux de la prospérité : plus de science pour créer des entreprises ; plus d’entreprises pour susciter de l’activité ; plus d’activité pour financer notre modèle social.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent texte vise non seulement à conforter le statut de la place financière de Paris, mais aussi à faciliter le financement des entreprises.

Sur le fond, notre première réserve porte sur l’article 1, qui autorise les entreprises à émettre des actions à droits de vote multiples lors de leur introduction en bourse. Le but est à l’évidence d’inciter certains entrepreneurs, notamment les dirigeants de PME innovantes, à se financer sur les marchés financiers tout en préservant le contrôle de leur société. Cette disposition doit être examinée à la lumière d’un exemple précis

Nos réserves auraient pu être plus fortes encore si les travaux accomplis en commission au Sénat n’avaient posé quelques garde fous – je pense notamment au maintien du principe « une action, une voix » pour les résolutions relatives à la rémunération des dirigeants et aux conventions réglementées. Notre deuxième réserve porte sur la possibilité, pour les fonds communs de placement à risques, d’accompagner les entreprises cotées jusqu’à une capitalisation boursière de 500 millions d’euros, contre 150 millions d’euros actuellement. Nous craignons qu’un tel choix ne favorise les entreprises de grande taille au détriment des start up.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Si le temps des réformes est souvent très long, il faut savoir se réjouir quand ces dernières voient le jour. C’est le cas aujourd’hui, avec la proposition de loi que nous nous apprêtons à examiner et dont nous ne pouvons qu’approuver les dispositions : elles améliorent la compétitivité financière de la France et facilitent le financement des entreprises par le marché.

Je pense, par exemple, à l’élargissement du champ d’investissement des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) aux marchés de croissance, comme Euronext Growth, dédiés aux PME et aux ETI innovantes ou encore à la simplification des règles d’éligibilité des titres des entreprises au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises, le PEA PME.

Seulement 12 % des PME comptent aujourd’hui un fonds d’investissement au capital de leur société. Notre modèle entrepreneurial reste fondé, en grande partie, sur l’actionnariat familial et se caractérise par le rôle prépondérant du secteur bancaire.

Nous devons avoir pour priorité de diversifier les sources de financement par les marchés financiers et le capital investissement tout en encourageant l’orientation de l’épargne vers les investissements dans les entreprises.

sont des entreprises familiales attachées à un territoire, à des salariés et à un projet de long terme. Mes chers collègues, le sommet Choose France est une bonne mais n’oublions pas les autres composantes de notre attractivité. Notre ambition doit aller au delà de ce texte : c’est une obligation morale envers tous les entrepreneurs, qui maintiennent la vitalité de nos territoires. La parole

proposition de loi n’est qu’un élément parmi d’autres pour – je répète son titre – « accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Compenser le déficit commercial de notre pays par le seul investissement financier est bien entendu une vue de l’esprit. De même, il est illusoire de croire que la seule dématérialisation de titres transférables

Nos entreprises ont soif de cotisations allégées, de formalités simplifiées, de formations et de ressources humaines adaptées. Sur tous ces points, notre pays a encore beaucoup de progrès à accomplir. Sait on qu’aujourd’hui

renferme en lui un risque de concentration du pouvoir entre les mains de quelques actionnaires qui, à l’aide de ce nouveau dispositif, pourront plus facilement s’assurer le contrôle de l’entreprise, avec le risque non négligeable que les détenteurs d’actions de préférence aient des motivations différentes

par la loi Pacte est une mesure récente dont les effets n’ont pas encore été évalués. Il serait donc opportun de mener une étude approfondie de cette mesure avant de l’étendre aux sociétés cotées en bourse – voilà encore une analyse dont l’absence d’étude d’impact nous prive. Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de supprimer l’article 1, dont les conséquences éventuelles sont manifestement mal évaluées et ne semblent répondre qu’à la fuite en avant de la concurrence entre les différentes places financières. Quel est l’avis de la commission des lois ? Cet amendement vise à supprimer

le développement de nos PME, risque d’avoir des conséquences néfastes sur leur pérennité. En effet, la financiarisation de ces dernières, c’est à dire la transformation d’entreprises ancrées dans l’économie réelle en véhicules financiers destinés à engendrer des profits pour les actionnaires, est une tendance dangereuse. En permettant la négociation de promesses d’actions sur les marchés, nous ne faisons qu’encourager cette dynamique. Par ailleurs, en assurant le coût du capital, notamment le paiement de dividendes aux actionnaires, les PME risquent de se retrouver sous une pression financière intenable. L’économie financiarisée et sa vision à court terme ont des conséquences sur l’emploi et le tissu économique local, puisque les PME ne sont

des salariés seraient alors mieux représentés au sein des conseils d’administration. En réservant cet outil financier à des acteurs présents dans la structure de l’entreprise, nous limiterions également le risque de prise de contrôle hostile par des investisseurs extérieurs, dont les intérêts pourraient diverger de ceux des employés ou des objectifs de long terme de l’entreprise.

Cet amendement est contraire à la position de la commission. Je le reconnais volontiers. Il vise à supprimer le plafonnement du ratio entre les droits de vote attachés aux actions de préférence et aux actions ordinaires sur les marchés réglementés.

Cette exclusion les prive d’un outil essentiel pour attirer les investisseurs, ce qui constitue un obstacle majeur à leur développement. Retenons que le dispositif proposé sera applicable aux SCIC qui prennent l’initiative de créer une réserve à cet effet.

car la loi ne le prescrit pas. C’est ce que nous proposons de changer. Il est temps de mettre un terme à la financiarisation de l’outil de travail des salariés sans les consulter à aucun moment, sous prétexte que les dirigeants seraient plus avisés. Nous suggérons donc une règle simple : si le comité social et économique (CSE) s’oppose à l’introduction en bourse,

puisqu’il s’agit de supprimer l’article 2, lequel prévoit d’élargir la possibilité pour les fonds communs de placement à risques d’accompagner les entreprises cotées jusqu’à une capitalisation boursière de 500 millions d’euros, contre 150 millions actuellement. Les FCPR bénéficient d’un traitement fiscal spécifique en cas de détention de titres pendant cinq ans. Ils permettent une exonération d’impôts sur les revenus et les plus values liés aux parts du fonds, si elles sont conservées pendant au moins cinq ans et si tous les revenus dans le fonds sont réinvestis pendant cette période. L’élargissement de l’éligibilité des FCPR soulève plusieurs inquiétudes. Premièrement, cela pourrait favoriser la croissance des FCPR existants au détriment de l’émergence de nouveaux acteurs, simplement par prédation, afin de leur permettre de bénéficier du régime fiscal spécifique. Deuxièmement,

8,32 milliards d’euros en 2023, pour un ticket moyen de 11,64 millions d’euros, bien loin des valorisations des entreprises cotées. Ce montant est en diminution de 38 % par rapport à 2022 et ne représente que les investissements sur le premier semestre de cette même année.

dont la plupart sont de toutes petites et moyennes entreprises non cotées, au mode de financement différent de celui des PME classiques et des entreprises cotées. Grâce à son cadre législatif incitatif, la France est

constitué d’une poche solidaire de 5 % à 10 % et distribué, entre autres, dans le cadre de l’épargne salariale et de l’assurance vie. Cet amendement tend notamment à porter le plafond de la poche solidaire à 15 %, sans modifier le plancher de 5 %. Cela permettra aux investisseurs

Comme avec l’amendement précédent, il s’agit de créer une incitation forte au financement des PME et des ETI en fléchant une partie des successions vers le financement de nos entreprises.

L’élargissement des critères risque de nous faire subir la critique de l’éviction telle que la subit aujourd’hui le PEA de droit commun. Pour ma part, j’aurais plutôt déposé des amendements allant dans le sens de la restriction des critères

entreprise solidaire d’utilité sociale », aujourd’hui uniquement attribué à des entreprises recherchant une utilité sociale. Son adoption risquerait de générer un effet d’éviction des financements actuellement fléchés vers des projets sociaux,

de considérer ses implications potentielles. Une augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription permet ainsi à l’entreprise d’ouvrir directement son capital à des tiers, sans que les actionnaires existants puissent souscrire à de nouvelles actions en priorité. Cela peut avoir un effet significatif sur la structure du capital de l’entreprise, sur sa gouvernance comme sur ses relations avec ses actionnaires. De plus, cette mesure pourrait susciter des réactions négatives sur les marchés financiers si elle était perçue comme une dilution des droits des actionnaires existants ou

Cet amendement vise à flécher 10 % d’augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne salariale.

monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cet amendement ayant déjà été discuté en commission, je prends naturellement en compte l’avis défavorable du rapporteur

La multiplication des informations communiquées aux autorités de régulation étrangères va mécaniquement entraîner une sollicitation supplémentaire de nos propres autorités, qu’il s’agisse de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou

aux impératifs de supervision financière et en aucun cas des informations de type industriel ou autres, qui mettraient en danger le secret des affaires. Je suggère donc de conserver cet article et de discuter du budget de l’Autorité des marchés financiers à l’occasion du projet de loi de finances, comme nous le faisons chaque

aujourd’hui. Il commence très fort : « Cocorico ! La France est le premier marché de la gestion d’actifs – c’est écrit en anglais dans l’article, mais nous sommes ici au Parlement français, nous parlons donc la langue de Molière – pour l’Europe continentale. Avec 4 589 milliards d’euros d’actifs sous gestion, l’Hexagone est loin devant la Suisse, l’Allemagne, les Pays Bas et l’Italie, d’après les derniers chiffres de l’association européenne de l’industrie de la gestion d’actifs, l’Efama. De quoi attiser les appétits de bien des maisons de gestion étrangères. étrangères. » Je crois que tout est dit. Pourquoi une telle mesure ? Pourquoi un tel intérêt des acteurs étrangers pour le marché français de l’épargne, considéré comme le premier marché d’Europe ? Il faut un associé du désormais célèbre cabinet de conseil McKinsey, cité dans le même article, pour rappeler que les équipes commerciales se tournent d’abord vers les acteurs institutionnels, mais que « les frais facturés sur les mandats, en particulier, sont très peu rémunérateurs. D’où l’appétence pour la clientèle individuelle qui, elle, ne représente que 30 % des volumes, mais 40 % des revenus.

de procéder à une offre au public de titres financiers, lorsque cette offre repose sur une infrastructure de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT), au sens du règlement européen sur le régime pilote La France a déjà adapté sa réglementation pour permettre aux SAS de participer au financement participatif, reconnaissant ainsi leur rôle essentiel dans l’économie. L’exclusion actuelle des SAS du régime pilote DLT va à l’encontre de cette tendance. Elle compromet les objectifs de l’Union européenne en matière d’innovation financière et de soutien aux PME. Je précise qu’il s’agit là d’une expérimentation. Il est question non pas de renverser la table,

Cet amendement vise à clarifier le régime d’émission des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, les BSPCE. Alors qu’ils sont attribués et qu’ils sont incessibles, car il ne s’agit pas de valeurs mobilières, le renvoi actuel au code de commerce est interprété par certains praticiens comme soumettant globalement les BSPCE au même régime que celui, contraignant, des valeurs mobilières. La charge administrative qui s’ensuit est d’autant plus lourde pour les émetteurs que les attributeurs de BSPCE sont larges, ce qui contrevient à l’objectif de favoriser l’actionnariat salarié. Le présent article vise donc à remplacer ce renvoi inopportun par une procédure d’émission classique, autorisée par l’assemblée générale extraordinaire, plus claire et source de sécurité juridique.

M. Michel Masset. Cet amendement vise à supprimer le doublon de contraintes administratives pesant sur les prestataires de services d’investissement (PSI) qui fournissent des activités de conseil en fusions acquisitions sur des sous jacents immobiliers,

de loi les entreprises qui ne prévoient pas l’indexation de leur salaire minimal conventionnel sur le Smic et qui délocalisent leurs activités à l’étranger.

engagements climatiques contraignants et à l’adoption de plans de « déplastification ». Nous souhaitons que toutes les entreprises bénéficiant des avantages prévus dans ce texte soient soumises à l’obligation de publier un bilan carbone complet, d’élaborer une stratégie climatique alignée sur une trajectoire de réduction des

des actionnaires. Une chercheuse en sciences de gestion expliquait voilà déjà une dizaine d’années que le vote par internet comportait « un inconvénient majeur en termes d’inégalité des actionnaires, car il n’existait pas de solution technique unique automatisant l’identification et facilitant la démarche de vote tous les actionnaires ». Elle faisait ainsi référence aux différences entre les actionnaires au porteur et les actionnaires non résidents, qui ne se trouvent pas dans les mêmes conditions, tout comme les actionnaires salariés, qui ne peuvent s’exprimer directement.

peut s’opposer à la tenue d’une assemblée générale en visioconférence. Nous proposons, par cet amendement, d’abaisser ce seuil à 5 %, l’objectif étant d’assurer l’effectivité de la démocratie d’entreprise.

Plusieurs solutions sont proposées, que je récapitulerai rapidement par souci de clarté. Certains entendent abaisser le seuil de capital social nécessaire permettant à un actionnaire de disposer de cette faculté, soit en fixant un nouveau seuil, soit en renvoyant à un décret qui fixerait le seuil. D’autres proposent de donner cette faculté à un groupe de 150 actionnaires au moins. Dans certains cas, toutes les sociétés sont visées, dans d’autres uniquement les sociétés cotées, dans d’autres encore celles dont le capital social est supérieur à 1 milliard d’euros.

force est de constater que le sujet n’entre pas véritablement dans les objectifs du texte que nous examinons ce soir, c’est à dire accroître l’attractivité de la France et, singulièrement, du droit français des sociétés. l’objet de l’amendement est assez éloigné de l’article 10, qui se limite à modifier le fonctionnement dématérialisé des organes sociaux. Enfin, d’autres questions plus fondamentales mériterait que l’on y consacre un travail spécifique en amont, mené en concertation avec les représentants des entreprises et des investisseurs. Il faut que nous soyons très prudents et que nous nous gardions de fixer des règles dont l’effet pratique pourrait être de complexifier inutilement le fonctionnement des sociétés. Nous savons par exemple que certains aux pratiques agressives utilisent l’arme des résolutions à la seule fin de déstabiliser le management, et nous serions mal avisés de faciliter cette tendance. Lors d’un débat similaire à l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’est engagé, en séance publique, à travailler sur la question du seuil et même à user, le cas échéant, des marges de manœuvre que lui donne son pouvoir réglementaire. Le ministre nous le confirmera peut être. Je vous propose de procéder par étapes. Dans l’attente de ces travaux, dont je pense qu’ils sont essentiels pour que nous ne manquions pas notre cible, j’ai proposé à la commission des lois de faire un premier pas en adoptant un amendement tendant à rendre plus efficaces les voies de recours juridictionnel des actionnaires minoritaires en cas de refus injustifié d’inscription à l’ordre du jour de résolutions qu’ils auraient proposées.

à favoriser la démocratie actionnariale en abaissant le seuil de détention de capital nécessaire au dépôt d’une résolution en assemblée générale, dans les grandes entreprises cotées en bourse, et en permettant à 150 actionnaires d’inscrire à l’ordre du jour des points ou des projets de résolution, indépendamment de leur part de capital.

En cas de rejet d’au moins l’une de ces deux résolutions, la rémunération variable et exceptionnelle des dirigeants de ces entreprises sera réduite de moitié. En donnant aux actionnaires plus de moyens pour évaluer la qualité des plans de transition des entreprises, c’est une nouvelle dynamique vertueuse orientée vers une finance plus durable

un avis défavorable

d’attirer des financements pour investir notamment dans les entreprises et la transition écologique. Le recours à des ordonnances se justifie par la technicité même des mesures concernées et par la nécessité d’échanges supplémentaires sur certaines dispositions et leur interaction entre elles, qui imposent de les considérer dans un ensemble cohérent.

puis transposé par le Gouvernement dans la loi : la question des FCPE de reprise a été abordée, mais pas les modifications que vous proposez. Au regard du consensus auquel sont parvenues les organisations syndicales et patronales, lequel a permis d’aboutir à cet accord, il me semble délicat de revenir sur ce sujet sans